l'amendement n° 330, qui vise à compléter la composition du conseil administration de France compétences à l'article 16. Cette composition figurant bien à l'article 16 du projet de loi, l'amendement tendait à prévoir des membres supplémentaires.

leur voie en toute connaissance de cause. Il s'agit donc d'offrir aux jeunes ayant des difficultés d'accès à l'apprentissage un dispositif les préparant à accéder à la formation et à intégrer le monde de l'entreprise. Ces actions seront comprises dans le seront comprises dans le programme national de l'État afin de répondre à un besoin additionnel de qualification au profit des jeunes sortis du système scolaire sans qualification. Quel est l'avis de la commission ?

et compagnons d'Emmaüs, travailleurs solidaires, développent les activités des communautés au sein desquelles ils vivent. Ces activités, souvent liées à la collecte d'objets, à leur réemploi, au recyclage et, plus récemment, à l'agriculture, développent une très importante solidarité à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Ces travailleurs solidaires que vous connaissez tous s'inscrivent dans des parcours d'insertion ou de réinsertion sociale. Il s'agit donc de dispositifs bénéfiques pour l'individu, mais aussi pour la société tout entière. Cette insertion sociale doit également être synonyme d'insertion professionnelle. C'est là tout l'objet du présent amendement. Les travailleurs solidaires pourront faire valoir une certification qualifiante auprès de leurs futurs employeurs et renforcer ainsi leur insertion professionnelle. Il s'agit, enfin, de faire inscrire dans la loi, la reconnaissance du travail des travailleurs solidaires et la promotion sociale que symbolise une VAE. Merci d'avance

toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ». Les travailleurs solidaires rentrent dans cette catégorie. À mon sens, les personnes visées par cet amendement sont déjà couvertes par le droit en vigueur. La commission a donc émis un avis défavorable.

La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l'article. L'article 5 du présent projet de loi porte sur l'évaluation de la qualité des formations professionnelles. Il ouvre notamment la possibilité que les formations soient évaluées par des « instances de labellisation Selon l'étude d'impact, la réforme du système de formation professionnelle vise à étendre les obligations de qualité à toutes les actions de formation et à harmoniser les pratiques afin de rendre le système de formation plus lisible. Dans ce but, vous avez annoncé, madame la ministre, vouloir aller « vers une certification des organismes », ce qui est une bonne chose. C'est d'ailleurs l'objet de l'article 5, qui prévoit que les formations seront évaluées par des organismes certificateurs accrédités. L'introduction d'une certification permet une meilleure lisibilité de l'offre de formation, à condition de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'organisme de certification. Or l'alinéa 7 de ce même article prévoit que les certifications peuvent être délivrées par les organismes certificateurs, mais également par des instances de labellisation. Ce terme ne fait référence à aucune structure existante et ne garantit nullement l'indépendance desdites instances à l'égard des organismes financeurs. Rien donc ne permet de s'assurer que les instances de labellisation accréditent les formations sur la base de critères objectifs, à part le référentiel national mentionné à l'alinéa suivant et dont on ne sait rien non plus, puisqu'il sera défini par décret. Il y a donc là un grand flou. Par ailleurs, l'instauration de deux instances distinctes chargées du même rôle de certification introduit, à notre avis, une inégalité entre les organismes formateurs, avec des actions de formation évaluées selon des modalités différentes.

Il vise plus particulièrement les établissements d'enseignement secondaire ou supérieur publics, les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'éducation et les établissements dont les formations sont évaluées par la commission mentionnée au même code. Il s'agit donc de mettre en place pour l'ensemble de ces établissements, qui dispensent également des formations par la voie de l'apprentissage, les mêmes règles que celles qui sont prévues pour les autres établissements.

associés à l'État par contrat dispensent des formations par voie d'apprentissage. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre de programmes et de référentiels nationaux fixés par le ministère de l'éducation nationale et élaborés par des procédures internes de validation. Les professeurs qui encadrent les élèves apprentis sont lauréats de concours de l'État dont le niveau d'exigence est élevé. Il apparaît donc inopportun et superflu de faire procéder à un contrôle supplémentaire par un organisme certificateur privé, alors que l'éducation nationale dispose en interne des ressources et procédures d'évaluation à partir de programmes et de référentiels validés par des procédures formelles. Il vous est donc proposé de supprimer l'alinéa 11.

l'Assemblée nationale à soumettre, avec l'accord du Gouvernement, les établissements secondaires publics et privés sous contrat à une obligation de certification qui vient s'ajouter aux contrôles que le ministère de l'éducation nationale est censé exercer sur ces mêmes établissements.

Le délai d'un an me paraît important. Il convient de rappeler que la certification exigée peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences, en l'espèce le ministre porteur du label qualité. Quel est maintenant l'avis de la commission

Cet amendement vise à permettre aux branches de compléter le pack minimum de critères de qualité fixés par décret dans la mesure où elles l'estiment nécessaire du fait de spécificités pouvant être liées à certains secteurs ou à certains métiers.

la commission ? Des règles existent actuellement pour assurer la qualité des formations dispensées dans les établissements concernés. Il ne me semble pas efficace de prévoir une conférence nationale de nature à introduire un formalisme et une bureaucratie inutiles. La commission émet un avis favorable.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, autorité administrative indépendante, évalue l'ensemble des établissements publics avant l'accréditation par le ministère, ainsi que les formations délivrées au nom de l'État. S'agissant des établissements privés, le Comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé procède à une évaluation complémentaire, après la première, afin de s'assurer de la participation au service public de l'enseignement supérieur des établissements qui bénéficient ensuite du label « établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général », ou EESPIG. S'agissant des écoles d'ingénieur, la formation conduisant au titre d'ingénieur diplômé par apprentissage requiert l'évaluation spécifique de la Commission des titres d'ingénieur. Toutefois, dans un souci d'amélioration continue de l'offre de formation, il est pertinent qu'une conférence annuelle réunisse tous ces acteurs et que France compétences puisse veiller non pas à l'accréditation elle-même ou à la labellisation, mais à la cohérence de l'ensemble des critères d'évaluation de la qualité des formations d'apprentissage.

concernant la pêche, tout marin doit, pour pouvoir naviguer, détenir des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les États signataires. Ces derniers sont également garants de la qualité des formations obligatoires délivrées en amont de l'acquisition de ces titres. Ces conventions imposent aux États signataires d'adopter un système interne de contrôle de la qualité de leur dispositif. fin, le code de l'éducation prévoit aujourd'hui, en son article R. 342-2, le principe d'un agrément des organismes délivrant des formations professionnelles maritimes, conformément à ces conventions, sans instaurer de sanction en cas de manquement de ces organismes. Cet article vise donc à rehausser au niveau de la loi ce principe tout en garantissant un strict respect de nos obligations internationales en matière de contrôle de la qualité des formations professionnelles maritimes. Dans un contexte où ce sujet fait souvent l'objet de polémiques, il est important

Le plan de formation est l'une des voies d'accès du salarié à la formation professionnelle continue ; il peut se faire à la demande de l'employeur ou à la demande du salarié. Actuellement, un salarié sur trois se forme. Si nous partageons la nécessité d'améliorer le système actuel pour permettre l'accès d'un plus grand nombre de salariés à des actions de formation professionnelle, le remplacement du plan de formation par un plan de développement des compétences nous semble être une régression pour les travailleuses et les travailleurs. Pour le Gouvernement, la formation professionnelle tout au long de la vie n'est plus l'occasion d'élargir les horizons des salariés, mais bien de les rendre le plus modulables modulables possible. Actuellement, les négociations collectives permettent de prendre en considération les besoins d'évolutions professionnelles des salariés dans les plans de formation. Demain, avec cet article, chaque salarié devra être capable d'anticiper les transitions économiques, écologiques et numériques, puisque la responsabilité de la formation, qui pesait sur l'employeur, pèse désormais sur l'employé. Lors des auditions par la commission des affaires sociales des organisations syndicales des salariés, le représentant de la CGT dénonçait l'absence de « réflexion sur la manière de réussir à bien faire son travail », soulignant que la « réforme renvoie la responsabilité de sa formation au salarié Cette déresponsabilisation des employeurs va de pair avec la formation des salariés en dehors des heures de travail. Certes, madame la ministre, ce n'est pas une nouveauté et le code du travail prévoit déjà une telle possibilité. Néanmoins, en déresponsabilisant les employeurs, vous allez mécaniquement augmenter le nombre d'actions de formation en dehors du temps de travail. Nous sommes profondément opposés au fait d'imposer aux salariés de choisir entre la formation professionnelle ou le temps de repos réservé à la vie familiale et sociale. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 6. Quel ? L'article 6 prévoit des avancées, notamment la fin de la distinction, relativement formelle et peu opérationnelle, entre les actions visant à l'adaptation et au maintien dans l'emploi et les actions de développement des compétences. Par ailleurs, je ne vois pas dans cet article les intentions que les auteurs de cet amendement prêtent au Gouvernement. La commission est donc défavorable

avoir un entretien au moment de l'embauche ainsi qu'au retour d'un certain nombre de congés : maternels, parentaux, sabbatiques, notamment. Cet entretien doit aussi être récurrent, car il a pour vocation de permettre à l'employé de faire le point sur ses perspectives d'évolution, d'emploi et de qualification.

d'une action de formation, d'une progression professionnelle ou salariale, ni de l'acquisition d'une certification quelconque. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale assouplit cette règle en prévoyant

même lorsque le salarié n'a bénéficié que de formations qui étaient obligatoires. Cela va à l'encontre de la logique qui est d'inciter les employeurs à développer les compétences de leurs salariés, par le biais de formations, au-delà du strict nécessaire. Par conséquent, la commission

possibilité de mobiliser son CPF pour suivre une action de formation coconstruite par le salarié et l'entreprise. ? Cet amendement est satisfait par l'alinéa 8 du présent article, dans la rédaction issue des travaux de la commission.

7 % des Français souffrent d'illettrisme, soit environ deux millions et demi de personnes, dont au moins la moitié travaille ; ils seraient plus nombreux dans l'industrie et en milieu rural. L'illettrisme est un phénomène difficile à cerner. Souvent, des stratégies de contournement sont développées par les personnes concernées pour ne pas avoir à se dévoiler. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme estimait que, plutôt que de transmettre des compétences techniques, qui seront rapidement obsolètes dans un environnement en perpétuelle mutation, il est nécessaire de conduire chaque individu vers la maîtrise d'un socle de compétences de base, vers l'autonomie et vers la capacité d'apprendre à apprendre, et de l'amener à s'adapter aux évolutions du travail, à pouvoir transmettre son savoir et acquérir de nouvelles compétences. C'est pourquoi nous estimons indispensable de conserver la mention des actions de formations spécifiques à la lutte contre l'illettrisme, et ce d'autant

d'actualiser leur dossier pour Pôle emploi ou leurs droits aux allocations familiales- on pourra dorénavant ajouter à ces actions inabordables du quotidien l'accès à la formation professionnelle un smartphone. Il s'agit là d'une nouvelle fracture sociale, qui concernerait un quart des Français. Le plan de compétences doit comporter une référence à la lutte contre l'illettrisme et au développement des compétences numériques, car, si l'entreprise n'y voit pas un intérêt économique immédiat- et encore -, il s'agit d'une exigence sociale et sociétale qui doit relever de la responsabilité de l'entreprise, dans un objectif d'émancipation de ses salariés. D'où cet amendement. commission ? L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et le maintien de leur employabilité. Il peut par ailleurs proposer des formations correspondant aux besoins de l'entreprise. Ainsi, les formations qu'il peut présenter à ses salariés sont très très nombreuses et diverses. En mentionner quelques-unes dans la loi ne me paraît pas pertinent, car cela pourrait être interprété comme une exclusion des autres. Je me permets de citer le rapport du Conseil d'État de 1991, qui constatait que, « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu'une oreille distraite De plus, il me semble évident que les formations concourant à la lutte contre l'illettrisme ou à la maîtrise du numérique correspondent tout à fait à l'obligation de maintenir une bonne employabilité. Donc l'employeur a même

Je suis un peu surpris de cette réaction. Notre réflexion et ce projet de loi portent sur la formation. L'ambition de ce texte est de faire que chaque salarié puisse s'épanouir et apporter à l'entreprise l'ensemble de ses qualités. Or il y a un élément fondamental, préalable à toute formation, quelle qu'elle soit : savoir lire et, aujourd'hui, savoir manipuler tous les outils électroniques qui sont utilisés. Celui qui ne dispose pas de ces atouts n'a aucune chance ... De la même façon que l'on définit les conditions dans lesquelles la formation peut se faire- les horaires, le financement -, une une autre condition est incontournable : celle de savoir lire et de savoir utiliser les nouveaux instruments. C'est pourquoi je trouve un peu étonnant que vous ne songiez pas,

Cela contrecarre le risque que les employeurs n'envoient leurs salariés en formation qu'en dehors de leurs heures de travail, afin d'éviter de réduire la capacité de production de l'entreprise ; mais cette limitation ne sera efficiente que s'il y a un véritable engagement des employeurs à libérer leurs salariés pour que ceux-ci suivent leurs formations.

que, par cohérence, le fait que ce ne soit pas une rémunération au sens de la sécurité sociale. Je vous ai entendue affirmer très fortement, tout à l'heure, qu'il faut renfoncer le droit à la formation ; d'accord, mais n'oubliez pas le droit social. Ainsi,

dit, cette mesure reflète une chose : les formations suivies en dehors du temps de travail ne sont plus considérées comme étant de la responsabilité de l'entreprise, quand bien même cette dernière en serait à l'initiative. Pourtant, les entreprises ont elles-mêmes tout intérêt à ce que les salariés suivent des formations. On peut donc s'interroger pourquoi un salarié sacrifierait-il son temps de repos pour suivre une formation de développement des compétences qui servirait en premier lieu à son employeur, surtout s'il n'a aucune contrepartie pour cet abandon de repos ?

est tout l'enjeu de cet amendement : permettre le maintien de l'allocation de formation qui doit servir à développer la formation des salariés, tout en assurant à ceux-ci des contreparties. En parallèle, cela doit permettre de rappeler la responsabilité des entreprises dans le processus de suivi des formations. Quel est l'avis de la commission ? Il est possible que l'alinéa visé par cet amendement soit erroné. En effet, l'alinéa 30 ne supprime pas cette allocation ; il modifie la dénomination du plan de formation, qui devient le « plan de développement des compétences Il pourrait être légitime de contester ce changement, mais il faudrait alors modifier chacune des occurrences, sous peine de créer une incohérence dans le texte. La commission émet donc un avis défavorable.

J'aurais souhaité une meilleure argumentation. On ne peut pas évoquer seulement un problème d'occurrences dans le texte

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, alors que nous entamons la discussion de l'article 7, qui simplifie les conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, je souhaite saluer l'esprit du projet de loi qui est, dès son intitulé, enthousiasmant projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, voilà un objectif que nous appelons tous de nos voeux, mais qui nécessite une réforme en profondeur de l'orientation. En réalité, de quoi parlons-nous ? De combattre les inégalités, en permettant à chaque élève de se réaliser vraiment dans la voie qui correspond à ses goûts, ce qui suppose de ne pas le conduire obstinément vers l'échec, souvent dans la voie que ses parents ont choisie pour lui, avec la complicité du chef d'établissement. Je rappelle que la France compte plus de 1,3 million de jeunes qui ne sont ni à l'école, ni à l'université, ni en apprentissage, ni dans la vie active. C'est un gâchis à la fois pour les jeunes, pour notre pays et pour l'économie. Parallèlement, de nombreuses entreprises artisanales peinent à recruter du personnel qualifié. Pourtant, nous le savons, l'apprentissage est l'un des meilleurs tremplins vers l'emploi. Alors, aborder la question de l'apprentissage dans un texte consacré plus largement à l'avenir professionnel peut paraître soit comme un premier pas vers une réforme plus profonde, soit comme bien trop réducteur, parce que le problème est avant tout un problème d'orientation dès le collège. Ce que je regrette également, c'est que la commission de la culture, de l'éducation et de la communication n'ait pas été saisie au fond, au même titre que la commission des affaires sociales, car le texte comporte plusieurs dispositions relatives à l'orientation scolaire, sujet sur lequel elle a beaucoup travaillé. L'apprentissage est un enjeu fort pour l'avenir de la jeunesse, parce qu'il est une voie d'excellence de formation aux métiers de l'artisanat et d'intégration dans l'entreprise,

Ces dernières semaines, le Gouvernement n'a cessé de dénoncer l'organisation actuelle et les chiffres de l'apprentissage, alors même que la dernière campagne fait état d'une hausse d'au moins 4,5 % du nombre de contrats, un record. Si nous partageons votre souhait de développer la voie de l'apprentissage, madame la ministre, nous ne pouvons vous suivre dans la voie de l'ouverture à la concurrence du marché de l'apprentissage. Cet article ajoute précisément l'insertion professionnelle parmi les objectifs assignés à l'apprentissage, et il remplace le dispositif d'enregistrement du contrat d'apprentissage, qui implique un contrôle préalable à son exécution, par une procédure de dépôt du contrat d'apprentissage auprès des futurs opérateurs de compétences, ou OPCO. Là aussi, si nous sommes favorables aux mesures de simplification, nous craignons que la suppression du contrôle du contrat d'apprentissage ne soit un mauvais signal envoyé aux apprentis quant à l'application de leurs droits- leurs droits- rémunération ou temps de travail, notamment. De même, nous ne partageons pas votre volonté d'éloigner l'apprentissage de la formation initiale pour l'orienter vers la formation continue. L'idée serait-elle de transformer, à terme, le contrat d'apprentissage en un contrat de professionnalisation ? La suppression de la référence à la jeunesse dans les objectifs et dans la définition de l'apprentissage fixés par la loi est symptomatique d'une volonté de diluer la spécificité de la filière. C'est la porte ouverte à l'augmentation de l'âge légal requis pour entrer en apprentissage, à laquelle nous nous opposons. Cela risque de déstabiliser le système et d'aboutir notamment à des contournements d'embauches en CDI, par le recours à des apprentis adultes à moindre coût. Il n'est pas inutile de rappeler que l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation et qu'il est, avant tout, une voie de formation pour les jeunes. Je regrette à mon tour

Lors de la discussion générale, j'ai indiqué que penser l'apprentissage dans le seul cadre du ministère du travail était une erreur, et que l'absence du ministère de l'éducation nationale limitait l'ampleur de la réforme. Or tout le monde en est d'accord, la rénovation de l'enseignement professionnel est une urgente nécessité. Développer d'abord l'apprentissage sans, en même temps, rénover la voie professionnelle, c'est mettre en danger les lycées professionnels, et mettre en place une loi visant à relancer l'apprentissage sans, en même temps, rénover la voie professionnelle, c'est s'inscrire dans un calendrier qui se déroulera aux dépens des lycées professionnels et de l'éducation nationale. C'est donc en même temps, madame la ministre, qu'il fallait construire une puissante rénovation de la voie professionnelle et de l'apprentissage et qu'il fallait, bien entendu, appuyer la rénovation de la voie professionnelle de l'éducation nationale sur une large utilisation de l'apprentissage et de l'alternance. C'est là que le « en même temps », aurait eu tout son sens. En lieu et place de tout cela, nous risquons au contraire d'avoir une relance partielle et cloisonnée et une rénovation de la voie professionnelle qui se fera, à tout le moins, sans passer par l'apprentissage ni par l'alternance. Malheureusement, la voie professionnelle et les lycées professionnels resteront donc les parents pauvres du ministère de l'éducation nationale.

apparemment, pas suffisamment pour que mes explications soient entendues. Je vous l'ai dit hier, mon collègue Jean-Michel Blanquer, ministre de l'éducation nationale, ma collègue Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et moi-même avons travaillé main dans la main

En parallèle, le ministre de l'éducation nationale a annoncé, voilà quelques semaines, une réforme des lycées professionnels qui va dans le même sens. Elle permettra une meilleure articulation entre l'apprentissage et le statut scolaire. Je pense qu'il est temps, en 2018, dans l'intérêt des jeunes de notre pays, de sortir de la querelle entre statut scolaire et apprentissage. Nous avons 1,3 million de jeunes qui cherchent leur voie ; il faut au contraire faire coopérer Qu'est-ce que cela signifie ? Que les lycées professionnels pourront tous ouvrir des sections d'apprentissage, je l'ai dit hier, et que, dans les campus des métiers, on favorisera aussi les passerelles entre statut scolaire et apprentissage, dans les deux sens- on pourra faire une partie de parcours sous une forme et une autre partie sous une autre. Ce sont deux voies pédagogiques : l'apprentissage, c'est « faire pour apprendre » et le statut scolaire, c'est « apprendre d'abord puis appliquer, faire ». Cela peut correspondre à des jeunes différents ou à des moments différents

prétendez, madame la ministre, vouloir développer et même revaloriser l'apprentissage, mais je crains que ce ne soit exactement le contraire qui se produise. Vous avez peut-être en tête, comme moi,

c'est précisément cela qu'il faut changer pour revaloriser l'apprentissage. Or, dans l'article 7, sont ouvertes des portes extrêmement inquiétantes ; cet article risque de faire de la voie de l'apprentissage non plus une voie de formation initiale, cela a été dit, mais une voie de formation professionnelle. Il risque de précariser encore un peu plus l'ensemble

sur le fait que l'apprentissage risque de devenir une nouvelle forme de salariat. Cela serait évidemment une nouvelle régression sociale. Voilà pourquoi nous proposons,

Elle facilitera ainsi pour les entreprises le recrutement d'apprentis. Par ailleurs, les entreprises pourront toujours être accompagnées et conseillées par les chambres consulaires, lors de la conclusion de contrats d'apprentissage. C'est pour cela que la commission émet un avis défavorable. Merci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

La commission a supprimé une disposition qui visait à confier la visite médicale d'embauche de l'apprenti à un professionnel de la médecine de ville, dans le respect des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article précité n'est disponible dans un délai de deux mois. Le motif en est qu'un médecin du travail connaît mieux le monde de l'entreprise qu'un professionnel de santé de la médecine de ville. Nul ne saurait le contester. Toutefois, il s'agit d'agir face à l'engorgement de la médecine du travail et de prendre en compte le fait que, sur le terrain, actuellement, les délais pour obtenir une visite médicale sont préjudiciables aux jeunes et aux chefs d'entreprise. Pour tenir compte de cette priorité que les apprentis doivent pouvoir rencontrer un professionnel de santé relativement tôt après leur embauche et afin de sécuriser l'entreprise au regard de ses obligations, le présent amendement tend, d'une part, à réintroduire la possibilité d'un recours à un professionnel de santé de la médecine de ville, dans le cas où un médecin du travail ne serait pas disponible dans les deux mois et, d'autre part, à préciser que, dans le cas où la visite d'information et de prévention est réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, la rémunération des apprentis concernés n'entre pas dans le calcul de la masse salariale déterminant la cotisation versée par l'employeur au service de santé au travail. de santé au travail. Ces amendements visent à rétablir la possibilité pour l'apprenti d'effectuer sa visite d'information et de prévention chez un médecin de ville si un médecin du travail n'est pas disponible dans les deux mois. La commission des affaires sociales a supprimé cette faculté. Elle a considéré que les apprentis, qui, bien souvent, découvrent le monde professionnel, ont besoin d'être conseillés par un médecin spécialiste du monde du travail, afin d'être sensibilisés aux risques auxquels ils peuvent être exposés.

Toutefois, cette gratuité n'exclut pas que les apprentis puissent payer une contribution pour financer des activités annexes à la formation, par exemple des activités culturelles et sportives de leur choix. C'est le cas de la contribution de vie étudiante et de campus, qui est due par les seuls étudiants, y compris les apprentis, des établissements de l'enseignement supérieur et des écoles de commerce, et qui sert à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants.

Nous estimons qu'un schéma satisfaisant consisterait à associer le groupement d'employeurs avec trois entreprises utilisatrices, dès lors que le groupement d'employeurs n'emploie pas réellement l'apprenti. Ce système permettra au groupement d'employeurs, donc aux très petites entreprises qui le composent, de faire appel à l'apprentissage, sans pour autant présenter pour eux un risque financier. n° 121. Je ne vais pas rappeler le rôle important des GEIQ dans nos territoires. Les GEIQ sont des structures à but non lucratif qui réunissent plusieurs entreprises dans l'objectif de qualifier et d'insérer des salariés dans la perspective de leur recrutement durable.

la mise à disposition dans le cadre des GEIQ est prévue et encadrée par le législateur et ne saurait être assimilée à un prêt de main-d'oeuvre illicite, même en cas de mise à disposition auprès de plusieurs entreprises, ce qui est d'ores et déjà le cas pour les embauches sous contrat de professionnalisation. L'objet de cet amendement est de favoriser l'apprentissage au sein des GEIQ, en permettant aux apprentis de bénéficier d'un cadre juridique ne limitant pas le nombre d'entreprises

Cette expérimentation peut être un levier de développement de l'apprentissage. En outre, limiter le nombre d'employeurs par apprenti à trois au sein d'un groupement paraît raisonnable, car un nombre trop important d'employeurs créerait des difficultés dans l'organisation de l'apprentissage et la cohérence de la formation.

L'objet de cet amendement est de définir une expérimentation relative à l'apprentissage pour les jeunes détenus jusqu'à 29 ans révolus, en tenant compte d'adaptations relatives à leur statut. Les conditions particulières seront précisées par décret. Tout le monde est conscient que la meilleure des préventions est la formation et l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, pendant la période d'incarcération, l'un des leviers essentiels de la réinsertion sociale des personnes condamnées est l'accès à l'emploi, à travers un d'activités : orientation et formation professionnelle, insertion par l'activité économique, insertion sociale et professionnelle des handicapés, travail au service général, en ateliers de production l'apprentissage peut s'inscrire dans cet objectif de favoriser la construction d'un parcours de détention orienté vers la préparation de la sortie. Les finalités du travail en détention sont d'inscrire les personnes détenues dans un processus de respect des règles, de concourir à leur équilibre par l'activité, de contribuer au maintien des liens sociaux et des relations avec le monde professionnel et de procurer une activité rémunératrice, qualifiante et valorisante qui prépare la sortie. Cet amendement vise donc à faciliter la réinsertion des jeunes détenus,

parce que tous les salariés auraient beaucoup à y perdre.

L'école doit favoriser la réussite de l'avenir professionnel. Pour cela, il convient de faire découvrir aux élèves de troisième et de quatrième différents grands secteurs professionnels, y compris ceux auxquels conduisent les lycées du même nom, ainsi que les formations en apprentissage Le but est de réduire, d'une part, le nombre bien trop important d'erreurs d'orientation lors du passage de seconde en première et, d'autre part, le nombre lui aussi bien trop grand d'élèves de terminale n'ayant aucun projet particulier pour les études post-baccalauréat. Cela passe par la création de passerelles entre écoles, entreprises, apprentissage et vie active. J'ai noté, madame la ministre, que ces passerelles étaient bien ancrées dans le projet par l'organisation, dès la classe de troisième, de véritables stages de découverte en entreprise, de découverte en entreprise, plus adaptés que ceux qui existent actuellement, et par une meilleure formation des enseignants sur les métiers. Les exemples de personnes ayant fait des études longues puis exercé un métier intellectuel pour ensuite devenir boulanger, cuisinier, menuisier ou agriculteur, par vocation, se multiplient aujourd'hui. Cette tendance indique clairement que rien ou presque n'est fait dans le cadre scolaire pour aider les jeunes à trouver leur voie. On sait, du reste, que nombre de métiers de l'artisanat souffrent d'un manque d'apprentis.

Faire découvrir les métiers de façon répétée est impératif. Cela doit se faire selon des modalités qui restent à déterminer pour les collégiens de quatrième afin de lutter contre de nombreuses erreurs d'orientation en seconde, comme contre l'absence de projet post-baccalauréat motivé chez un nombre trop important d'élèves de terminale.

Seront ainsi évoqués la hausse de la limite d'âge de l'entrée en apprentissage, à 29 ans révolus, la modulation de la durée du contrat d'apprentissage, l'allongement de la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire des apprentis, y compris mineurs. L'article 8 traduit un affaiblissement des protections des apprentis. Il constitue une dérégulation du droit du travail s'appliquant en matière d'apprentissage, au service des besoins immédiats et locaux des entreprises. Des possibilités de commencer un apprentissage ou une formation en alternance au-delà de 25 ans existent déjà lorsque certaines conditions le justifient. On nous parle souvent de ces jeunes adultes qui découvrent tardivement leur voie et ont envie de vivre leur passion.

ni de savoir-être concrets. L'article 8 est plutôt une invitation à contractualiser sur des critères flous, comme le niveau initial ou les compétences requises. Cette situation est évidemment défavorable à l'apprenti, souvent jeune et pas toujours en capacité de négocier les termes de son contrat.

Cet article prévoit également d'assouplir la réglementation applicable à la durée de travail hebdomadaire, ce qui est en soi une bonne chose. Cela permettra d'adapter l'entrée en apprentissage et les métiers de l'apprentissage aux besoins réels et concrets du terrain et des différents secteurs.

dit, ces évolutions vont dans le sens d'une plus grande adaptation de la société aux évolutions du marché du travail et des spécificités des différents secteurs et des différentes branches. Je voudrais évoquer deux points

Depuis la première mention d'un âge d'instruction obligatoire, en 1882, l'ensemble des réformes a visé à allonger ce temps de scolarisation pour arriver, depuis 1959, à une fourchette de 6 à 16 ans. De fait, en

1970. À la fin des années 2000, un nouveau phénomène de contournement de la période d'instruction obligatoire est apparu. Nous pensons, bien évidemment, à la formation d'« apprentis juniors », instaurée par la loi de 2009, aux écoles de production, que certains réintroduisent texte après texte, ou aux dispositifs de préapprentissage. Ces derniers posent des problèmes de plusieurs ordres : on peut s'interroger sur l'honnêteté de ces cursus qui, tout en permettant de respecter la loi en conservant un statut scolaire, ne sont déjà plus de la scolarisation, mais de la préparation opérationnelle à un emploi. Il s'agit ensuite

Enfin, ces dispositifs de professionnalisation précoce sont trop souvent une solution de facilité pour mettre de côté des jeunes fréquemment en difficulté. Gouvernement après gouvernement, plutôt que de réunir les conditions pour amener tous les élèves à un niveau de connaissance suffisant leur permettant de s'émanciper des contraintes sociales et d'appréhender au mieux le monde dans lequel ils évoluent, on préfère, dès le plus jeune âge, enfermer des adolescents dans des parcours professionnalisants, à la formation disciplinaire limitée. jeunes sont capables, à 13 ou à 14 ans, de s'inscrire réellement dans un parcours professionnel abstrait ? C'est pour ces trois raisons que nous souhaitons revenir à une professionnalisation démarrant réellement à 16 ans, à la fin de l'instruction obligatoire. Il s'agit ici du schéma logique de l'instruction en deux phases : une période obligatoire assurant à toutes et à tous un enseignement suffisant pour réfléchir sereinement à son orientation, puis une période plus progressive au cours de laquelle l'orientation ne se fait plus par l'échec, mais par une construction du projet professionnel. L'amendement

Cet amendement vise à revenir sur l'allongement de la durée légale du travail des apprentis. L'article 8 de ce projet de loi permet aux entreprises de déroger à la durée légale du travail et de faire travailler les apprentis jusqu'à dix heures par jour et quarante heures par semaine lorsque l'organisation collective du travail le justifie. Il faut tout d'abord rappeler que l'apprentissage est ouvert dès l'âge de 16 ans et qu'il concerne majoritairement des jeunes ayant entre 16 et 20 ans, comme le souligne un rapport du ministère de l'éducation nationale de 2017. À ce titre, les apprentis doivent bénéficier de règles spécifiques tenant compte de leur âge et de leur condition physique. Ensuite, faire travailler les apprentis un aussi grand nombre d'heures et leur faire suivre l'horaire collectif revient à les traiter comme les autres salariés. Or le but de l'apprentissage est avant tout d'offrir une formation et de transmettre des compétences aux apprentis, non de fournir aux entreprises une main-d'oeuvre au rabais non seulement les apprentis ne devraient pas pouvoir travailler au-delà de la durée légale, mais leur temps de travail devrait être limité à six heures et demie Une telle disposition permettrait de préserver les plus jeunes et d'offrir à tous le temps nécessaire pour suivre correctement leur formation théorique.

Il existe un salaire minimum légal pour chaque tranche d'âge qui correspond à un pourcentage du SMIC en vigueur au 1 janvier. Ainsi, selon le site du service public, le salaire minimal d'un apprenti en première année est de 25 % du SMIC, 372 euros, s'il est âgé de 15 à 17 ans ; de 41 % du SMIC, soit 614 euros, entre 18 et 20 ans ; à partir de 21 ans, 53 % du SMIC, soit 794 euros. Un apprenti en deuxième année verra son salaire légèrement progresser. En troisième année, les apprentis les plus âgés, c'est-à-dire 30 ans avec ce texte, gagneront au maximum 78 % du SMIC, soit 1 168 euros. Sous prétexte que les différences de salaires selon l'âge conduisent à une inégalité entre apprentis d'une même année d'études, vous proposez d'uniformiser vers le bas cette échelle des salaires. Pour

de débuter un apprentissage s'il a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ou une « prépa métiers ». Supprimer cette dérogation défavoriserait les jeunes nés en fin d'année ayant terminé leur scolarité au collège et souhaitant débuter un apprentissage sans pouvoir signer de contrat, faute d'avoir atteint, à quelques semaines ou à un mois près, l'âge de 16 ans.

L'article 8 prévoit au contraire que les apprentis pourront, dans certains secteurs, travailler jusqu'à dix heures par jour et quarante heures par semaine, en bénéficiant de repos compensateurs. Ces dérogations permettront aux apprentis de s'adapter au rythme de travail de l'entreprise dans un grand nombre de secteurs soumis à des contraintes horaires, en particulier dans l'artisanat, l'hôtellerie ou encore la restauration. Elles faciliteront l'embauche et l'intégration des apprentis

passent du temps à les former correctement plutôt qu'à leur demander une production. C'est d'ailleurs ce qui se fait dans tous les métiers. J'ai moi-même été maître d'apprentissage pendant ans. Si la loi fixe un minimum en pourcentage du SMIC, la rémunération de l'apprenti peut être plus favorable au bénéfice de dispositions contractuelles ou conventionnelles. C'est d'ailleurs très souvent le cas dans l'enseignement supérieur. Pour ces raisons, la commission est défavorable

Vous autorisez ainsi le basculement de l'apprentissage vers la formation continue et fragilisez l'accès des plus jeunes à l'apprentissage, et ce

quel fondement ? Selon nous, il convient, à tout le moins, de laisser cette expérimentation aller jusqu'à son terme et d'établir une réelle évaluation de laquelle devra découler une généralisation ou un arrêt, selon les résultats avérés.

Après cette année d'expérimentation, les acteurs de l'apprentissage auditionnés par vos rapporteurs accueillent favorablement cette généralisation de l'entrée en apprentissage jusqu'à 29 ans révolus qui ne remettra pas en cause l'apprentissage en tant que formation professionnelle initiale. Ce rehaussement de la limite d'âge se combine utilement avec les possibilités d'effectuer un apprentissage pour une période de six mois minimum et de prendre en compte les acquis préalables de l'apprenti pour moduler la durée de sa formation.

des connaissances et d'apprendre un métier, mais il ne doit pas être que cela. Il faut aussi que les candidats à l'apprentissage en sortent avec des compétences théoriques qui leur permettront de continuer à exercer plus tard des métiers peut-être différents, à tout le moins de s'insérer durablement

de la commission ? Le droit en vigueur permet déjà d'effectuer un apprentissage compris entre six mois et un an, notamment lorsque l'apprenti prépare un diplôme d'un niveau inférieur à un diplôme déjà obtenu ou lorsqu'il a validé des compétences par la VAE, La généralisation de la durée minimum de six mois est donc de nature à développer l'apprentissage. Elle est utile pour tenir compte des acquis préalables de l'apprenti ou encore dans le cadre de réorientations professionnelles. Quand on choisit

permet à un jeune de suivre normalement sa formation en CFA pendant un an, même s'il n'a pas trouvé d'employeur. Cela pose des problèmes en fonction de l'aménagement du territoire, comme vous le savez. Beaucoup de jeunes renoncent à l'apprentissage, faute d'avoir trouvé un maître d'apprentissage. La mesure que nous souhaitons rétablir permet d'éviter, dans cette situation, que le jeune ne

dans la même entreprise afin de rendre le dispositif plus opérationnel et plus souple. En outre, avoir la possibilité de faire plusieurs stages organisés par le CFA dans la même entreprise pendant cette année d'aménagement particulier du cursus est susceptible de favoriser la conclusion d'un contrat d'apprentissage avec ladite entreprise. Quel

du syndicat de leur choix afin de faire valoir leurs droits dans les dispositifs de médiation que vous souhaitez instaurer en matière de rupture du contrat d'apprentissage. Quel est l'avis de Le droit du travail garantit déjà à tout salarié l'exercice du droit syndical et du droit de grève. Ces droits sont donc déjà garantis aux apprentis et cette précision n'est pas nécessaire. En outre, le code du travail prévoit que le délégué syndical doit être âgé de 18 ans révolus. Il ne serait pas très opportun qu'un apprenti représente les salariés de l'entreprise, compte tenu de son statut particulier. La commission a donc émis un avis défavorable

Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, technologique et pratique en vue d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique, voire un titre d'ingénieur ou un titre répertorié. La possibilité d'allonger la durée maximale de travail des apprentis rompt l'équilibre entre le temps de travail, le temps d'études et le temps de repos. Or cet équilibre est plus que nécessaire : l'apprenti n'est pas un travailleur comme les autres, c'est avant tout un jeune en formation qui a besoin d'un régime protecteur. La loi actuelle prévoit déjà des dérogations pour certains métiers : les dérogations accordées par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement. Il n'est donc nul besoin d'élargir encore ces dérogations, d'autant plus que les alinéas mentionnés dans le présent amendement concernent aussi les jeunes mineurs.

qui vise à ne pas limiter le repos compensateur des heures effectuées en dépassement des durées maximales au seul dépassement de la durée quotidienne, mais de le prévoir pour tout dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire. L'amendement n° 300, présenté par Mme Féret,

Ces garanties s'accompagneront de repos compensateurs. Ces mesures permettront aux apprentis de s'adapter au rythme de travail de l'entreprise dans un grand nombre de secteurs soumis à des contraintes horaires. Elles faciliteront l'embauche et l'intégration est défavorable à l'amendement n° 296. Les dispositions de l'amendement n° 300 sont cohérentes avec la position de la commission sur la médecine de ville : un médecin du travail sera mieux à même d'apprécier si un dépassement exceptionnel de la durée maximale hebdomadaire

dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, d'exécuter le contrat d'apprentissage en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique Je propose d'étendre cette disposition aux collectivités du Pacifique qui devraient, elles aussi, pouvoir bénéficier d'un renforcement des échanges avec les territoires du voisinage du même bassin océanique. La situation de l'emploi des jeunes dans les outre-mer est très préoccupante. En Nouvelle-Calédonie, le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans s'élève à 36 %. La généralisation des mobilités des apprentis ultramarins vers les pays d'Europe n'est pas en raison des difficultés d'adaptation de nos jeunes et du coût élevé des déplacements. Ainsi, il serait plus judicieux de favoriser les déplacements des apprentis à l'étranger, dans leur environnement géographique propre.

prévoit que les apprentis pourront aussi bien effectuer une mobilité à l'étranger, dans l'Union européenne ou à l'extérieur de l'Union européenne.

ainsi proposé de compléter les dispositions du code du travail relatives au mode d'apprentissage, en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles dont l'adéquation des compétences avec la formation aura été vérifiée.

Une telle mesure permettra en effet de développer l'apprentissage dans le secteur associatif. S'ils poursuivent les mêmes objectifs et doivent avoir les mêmes effets, ces amendements n'ont pas exactement la même rédaction.

pénale ? C'est une piste dangereuse ! Le sujet a été réglé dans le domaine des associations sportives par la législation, qui reconnaît le dirigeant du club sportif comme employeur.

pour garantir l'accomplissement et la réussite du contrat d'apprentissage. C'est pourquoi une formation pédagogique certifiante obligatoire nous paraît indispensable. Cette exigence de formation pédagogique permettra en outre de lutter contre les ruptures prématurées de contrats d'apprentissage,

bénéficie des formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti. L'article 19 précise que les opérateurs de compétences prendront en charge les actions de formation pour les maîtres d'apprentissage. Ajouter une obligation supplémentaire de formation certifiante

de l'apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme préparé, quel que soit son âge. Aujourd'hui, la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation, ce qui nuit à l'embauche des apprentis plus âgés. À diplôme et niveau de formation égaux, la rémunération d'un apprenti majeur est plus élevée que celle d'un apprenti mineur. Alors même que les candidats à l'apprentissage provenant d'une réorientation, souvent post-bac, sont en augmentation - 30 % des candidats entrés en apprentissage en 2015-2016 sont dans ce cas

? Dans les faits, les apprentis passent en général la majeure partie de leur apprentissage en entreprise. Il est en effet préférable que la formation pratique soit prépondérante. Toutefois, indiquer que le temps en entreprise est prépondérant risquerait de figer dans la loi une organisation, qui, à l'heure actuelle, permet aux apprentis d'acquérir une formation pratique sur les plateaux techniques des CFA

en adaptant les parcours ; d'un autre côté, Mme la ministre s'apprête à supprimer le dispositif des stagiaires de la formation professionnelle. Vous le savez, celui-ci vise à assurer une formation à des jeunes qui souhaiteraient suivre un cursus en apprentissage, mais n'auraient pas trouvé d'entreprise. Concrètement, ces jeunes s'inscrivent en CFA et sont autorisés à y suivre les cours durant un an. Ce dispositif a - ou avait ! - deux intérêts majeurs. Premièrement, évite le déclassement de ces jeunes, qui, sinon, se retrouveraient sans formation et sans emploi. Deuxièmement, il peut aussi représenter une opportunité lorsque l'on n'est pas sûr de son projet professionnel, grâce à la multiplication des expériences en entreprise.

chose. Nous l'avons souligné au cours du débat, il est de plus en plus difficile pour les apprentis de trouver des entreprises où effectuer leur apprentissage. On

Le scrutin est ouvert.

En effet, selon une enquête de la chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France de 2016, plus de 20 % des patrons de TPE et de PME refusent de recruter un apprenti, car ils estiment ne pas pouvoir le confier à un encadrant. Il est vrai qu'être chargé de former un jeune à son travail sur des périodes continues plus ou moins courtes représente forcément une responsabilité, donc une charge. De fait, cela demande un investissement en temps important, parfois incompatible avec les propres tâches du salarié encadrant. Cet amendement prévoit donc que le maître d'apprentissage bénéficie d'avantages en rémunération ou en jours de repos. L'enjeu est bien de motiver les salariés à assumer cette tâche. Concrètement, la disposition vise à laisser aux branches le soin de définir la formule la mieux adaptée : une prime ou un repos compensatoire. Il me semble que, sur ce sujet, beaucoup de choses pourraient être faites. L'introduction d'une valorisation est un premier pas pour rendre attractive la charge d'un suivi d'apprenti. Car, mathématiquement, si l'employeur doit, en vertu du code du travail, permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail des moments d'accompagnement d'un apprenti, il faut bien trouver une solution pour que le travail soit effectué. Et bien Et bien souvent- vous le savez, mes chers collègues -, c'est des heures supplémentaires que le maître d'apprentissage arrive à remplir toutes ses obligations. C'est tout l'enjeu du mécanisme de repos compensatoire que d'accorder aux maîtres d'apprentissage une compensation à leur investissement jusqu'ici purement bénévole. Quel purement bénévole. Quel est l'avis de la commission ? Une gratification pour les maîtres d'apprentissage risque d'inciter à l'exercice de cette fonction pour des raisons financières et de freiner l'embauche d'apprentis par les entreprises il faut laisser l'employeur libre de ce genre d'initiative. En outre, le code du travail prévoit déjà que l'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.

54 % des jeunes interrogés considèrent que les apprentis n'ont pas de bonnes conditions de travail. Cette opinion n'est pas contrebalancée par le niveau de la rémunération, puisque seuls 18 % des jeunes considèrent que les apprentis sont bien payés, 70 % d'entre eux affirmant le contraire. Seuls 12 % des jeunes sondés affirment que les apprentis ont facilement accès à un logement ; ils sont 58,7 % à penser le contraire.

Le coût des trajets entre le domicile et le lieu de travail réduit d'autant le montant des salaires des apprentis. Nous proposons donc que, dans les entreprises de plus de onze salariés, l'employeur prenne à sa charge la moitié des frais de transport personnels de l'apprenti, tout en précisant que cette prise en charge ne peut être déduite du salaire de l'apprenti. Quel Les entreprises prennent déjà en charge les frais de transport des apprentis, au même titre que ceux des salariés. Accroître la contribution des entreprises au financement des frais de transport risque de freiner le recrutement d'apprentis.

des publics jeunes, qui font très tôt le choix de l'apprentissage, des publics pour lesquels le code du travail apparaît obscur et flou, et qui ignorent jusqu'à leurs droits. Ces publics ont un besoin urgent d'accompagnement ; il convient de leur apporter les réponses

si le travail est bien fait, ce que vous proposez doit déjà être prévu. En effet, la loi dispose que l'apprentissage concourt au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté. les enseignements dispensés dans les CFA, qu'ils soient théoriques ou qu'ils aient lieu sur des plateaux techniques, doivent permettre aux apprentis d'acquérir un savoir-être en milieu professionnel. En la matière, d'apprentissage a aussi un rôle prépondérant à jouer : il est en quelque sorte le tuteur de l'apprenti. Il n'apparaît donc pas nécessaire de figer cette obligation dans la loi en créant des contraintes sur les bénéficiaires et sur la durée d'un tel module. Une telle obligation serait une charge supplémentaire à ajouter au coût de l'apprentissage. Quel est

les classes « prépa-métiers », qui constituent à nos yeux un détournement de l'obligation d'instruction jusqu'à 16 ans. Comme le montrait, en septembre 2016, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, et comme le montrent aussi de multiples études, l'école républicaine ne joue pas son rôle d'ascenseur social et ne contribue pas à résorber les inégalités sociales : elle contribue même à les creuser.

Son remplacement par une troisième « prépa-métiers » apparaît donc intéressant en vue de préparer des jeunes à la voie professionnelle tout en les maintenant au collège, où ils recevront le même socle de connaissances que les autres élèves.

cas dans le cadre de la loi de 2011, afin de préparer le plus en amont possible l'orientation de ces élèves et leurs perspectives professionnelles. Il ne s'agit pas d'enfermer des jeunes

par des enseignements dédiés et des stages, sans renoncer à la transmission du socle de connaissances prévu pour ces élèves. Nous avons des doutes sur la portée de ce dispositif et sur son articulation avec les « prépa-pro » qui existent au collège. Préparer des élèves de quatrième, 13 ou 14 ans, à la voie professionnelle nécessiterait des aménagements par voie réglementaire, notamment pour que le temps de stage soit progressif de la quatrième à la troisième.

prêts à se remobiliser autour d'un projet de formation, un accompagnement dans la construction d'un projet vers la voie professionnelle et l'apprentissage ; cette classe permet de renforcer la découverte des métiers tout en poursuivant l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Mais la création de la prépa-métiers n'a pas pour objectif de créer des filières dès la classe de quatrième ; le risque, bien réel, serait, pour le jeune, de ne plus pouvoir repartir vers d'autres voies. Il faut qu'à tout moment le jeune ait le choix.

dispositif aux élèves de quatrième pourrait nuire à l'acquisition des éléments fondamentaux qui constituent le socle commun nécessaire à la mobilité professionnelle. Qu'il y ait besoin d'agir, en matière de prévention du décrochage scolaire,

aux contraintes du système. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est un secteur d'activité en tension où les difficultés de recrutement sont très fortes et deviennent un véritable problème, en particulier dans les zones les plus touristiques de notre pays, dont on souhaite qu'il demeure la première destination touristique mondiale. Afin d'accroître le nombre de candidats potentiels à l'intégration d'une filière d'apprentissage dans le secteur de la restauration, il est proposé d'ouvrir cette possibilité à tous les mineurs dans les conditions de droit commun, soit, selon les termes de l'article L. 6222-1 du code du travail, à partir de 16 ans ou dès 15 ans pour les mineurs qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Cela éviterait de laisser au bord du chemin les jeunes qui ont terminé leur scolarité de premier cycle et qui souhaitent s'engager dans une filière professionnelle fortement pourvoyeuse d'emplois dans des zones géographiques attractives. Les dispositions proposées garantissent en outre la coordination de cette nouvelle rédaction du code du travail avec l'article correspondant dans le code de la santé publique.

des anciens CAP « Employés de restaurant », « Service en café-brasserie » et « Service hôtelier », est source de nombreuses difficultés pour les jeunes de moins de 16 ans, qui ne sont plus autorisés à souscrire un contrat d'apprentissage en vue de préparer ce nouveau CAP. À ces jeunes, il est opposé une fin de non-recevoir quant à la possibilité de suivre une formation dans un domaine qu'ils ont au préalable choisi en connaissance de cause, et pour lequel ils se sont pleinement engagés. C'est peu compréhensible eu égard à l'esprit de simplification qui anime le Gouvernement, et à l'heure où ce dernier annonce faire du développement de l'apprentissage une de ses priorités. En effet, aujourd'hui, nombre de jeunes sortant de troisième, et donc éligibles à l'apprentissage et/ou aux stages, ont, du fait d'un faible taux de redoublement, moins de 16 ans, voire 15 ans. Cet amendement vise donc à ouvrir cette possibilité d'apprentissage à tous les mineurs à partir de 16 ans, ou dès 15 ans pour ceux qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

telle extension s'inscrit dans la logique de l'article 8 , qui vise à faciliter l'emploi d'apprentis dans les entreprises de débit de boissons, comme les cafés, hôtels et restaurants. Cela permettra aux apprentis de 15 ans ayant validé leur scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire de bénéficier des mêmes dérogations que les apprentis mineurs d'au moins 16 ans.

Cet amendement a pour objet de supprimer la disposition facilitant les modalités de rupture du contrat d'apprentissage. Cet article crée en effet de nouveaux cas de résiliation unilatérale du contrat sur l'initiative de l'employeur et prive les apprentis de la protection des conseils de prud'hommes. Actuellement, un employeur qui souhaite mettre fin au contrat de son apprenti peut librement le faire pendant les quarante-cinq premiers jours. Au-delà de ce délai, sauf accord des deux parties, la rupture du contrat ne peut être prononcée que par un juge. Cette protection particulière de l'apprenti se justifie notamment par le fait qu'il n'est pas un salarié comme les autres. Il s'agit d'un salarié en formation. L'employeur qui l'embauche prend la responsabilité de le former et ne doit pas pouvoir mettre fin à son engagement sans sans contrôle, d'autant plus que la rupture du contrat de travail de l'apprenti met bien souvent fin à sa formation, l'empêchant d'obtenir son diplôme. Cet article fait référence à un médiateur rattaché aux tribunaux de commerce. Il est déjà possible pour une entreprise et son apprenti d'avoir recours à un médiateur lorsqu'ils ont la volonté de résoudre un différend. Or, bien souvent, lorsque l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat d'apprentissage, c'est qu'il est déjà trop tard pour résoudre le différend. C'est pourquoi, en cas de rupture du contrat, l'intervention d'un médiateur ne doit pas pouvoir remplacer celle Enfin, pour rappel, le taux de rupture des contrats d'apprentissage s'élève actuellement à 27 %. Il apparaît paradoxal que cette loi prétende prétende favoriser l'apprentissage tout en facilitant les ruptures de contrat, ce qui aurait pour conséquence inévitable d'augmenter le nombre d'apprentis n'ayant pas pu achever leur formation. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

! L'article 9 assouplit les conditions de rupture du contrat d'apprentissage tout en maintenant des garanties pour l'apprenti : rapprochement avec les conditions de rupture d'un contrat à durée indéterminée et intervention du médiateur consulaire.

Gay. Cet amendement a pour objet de lutter contre un des fléaux de l'apprentissage : le nombre de ruptures de contrat. Plus d'un quart des contrats signés sont rompus avant leur terme, dans un cursus qui est souvent vu comme le dernier rempart contre le déclassement.

au cours du cursus, c'est bien souvent particulièrement difficile pour ces jeunes apprentis. Il faut se mettre à leur place : soit l'apprentissage relève d'un choix propre, et c'est tout un plan d'avenir qui s'effondre soit ils ont été poussés vers cette voie trop souvent dévalorisée, et la déclaration d'inaptitude constitue la fermeture de la dernière porte pour obtenir une qualification. De la même manière, il s'agit aussi bien souvent d'un moment difficile pour les employeurs, qui, d'une part, ont souvent construit leur équipe avec l'apprenti et, d'autre part, se sont engagés. Le dispositif que nous proposons consiste à prévoir un reclassement pour inaptitude qui permette à la fois aux jeunes de voir leur réorientation facilitée et aux employeurs d'avoir une certaine stabilité dans leur effectif. On peut par exemple penser aux allergies qui se déclenchent parfois à l'âge adulte, notamment vis-à-vis des matières premières. Par exemple, un apprenti boulanger qui commencerait à souffrir d'une allergie à la farine pourrait changer de métier tout en restant dans la même structure, en s'orientant vers l'aspect commercial de l'entreprise. Bien entendu- c'est un élément à prendre en compte -, on parle de jeunes qui voient leur plan d'avenir remis en cause ; cela implique une certaine pédagogie et un accompagnement dans la réorientation.

Cette proposition est contraire à l'objectif de l'apprentissage. Si l'apprenti est inapte à occuper le poste correspondant au métier qu'il a choisi et prépare par l'apprentissage, son reclassement à un autre poste dans l'entreprise, qui est très souvent une petite entreprise, relève tout simplement de l'utopie.

loi. La loi du 5 mars 2014 a apporté une réforme majeure en matière de résiliation du contrat d'apprentissage, puisqu'elle permet d'obtenir rapidement une décision en matière de rupture du contrat, en donnant compétence au conseil des prud'hommes qui statue en la forme des référés. Dans l'étude d'impact, les raisons pour lesquelles une telle évolution est proposée ne sont pas spécifiées. Aucun chiffre ne permet de savoir ce qu'il en est de l'efficience de la procédure ouverte voilà un peu plus de quatre

: La parole est à Mme Pascale Gruny. La force majeure doit être prévue comme mode de rupture par anticipation du contrat d'apprentissage, comme elle est prévue dans le cadre du CDD ou du contrat de travail temporaire.

sur l'intervention du médiateur. La phrase retenue est très énigmatique alors que les chefs d'entreprise ont besoin de dispositions claires. Tel que l'alinéa est rédigé, l'intervention du médiateur semble constituer une obligation avant un licenciement,

La parole est à Mme Nathalie Delattre. Actuellement, de simples difficultés économiques de l'entreprise ne sont pas considérées par le juge comme un motif de résiliation du contrat d'apprentissage. Seule la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de l'entreprise autorise la rupture anticipée. Aussi, notre amendement prévoit une possibilité de rupture du contrat de l'apprenti en cas de difficultés économiques de l'entreprise. Il serait en effet préjudiciable de poursuivre l'exécution d'un contrat d'apprentissage dès lors que l'activité ne permet pas d'offrir à l'apprenti des conditions de formation

Actuellement, une rupture anticipée du contrat d'apprentissage motivée par la dégradation de la situation économique de l'entreprise ne peut intervenir qu'en cas de liquidation judiciaire, sur décision du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce. Il serait utile de permettre aux entreprises

afin de ne pas décourager l'embauche d'apprentis dans un contexte économique dégradé, en prenant notamment en compte le manque de visibilité financière des TPE au moment de au moment de l'embauche de l'apprenti. Il s'agit également d'éviter, en cas de difficultés économiques sérieuses rencontrées par l'entreprise, de contribuer à la dégradation de sa situation financière, en poursuivant l'exécution d'un contrat d'apprentissage, alors même que l'activité réalisée ne permet plus d'offrir à l'apprenti des conditions de formation satisfaisantes. L'intervention préalable du médiateur serait évidemment nécessaire.

du contrat d'apprentissage. On remarquera en effet que rien n'est prévu en la matière, ce qui est source d'insécurité juridique. Ces dispositions s'inspirent de celles de l'article L. 1243-5 du code du travail dans le cadre du CDD.

la commission ? Le passage obligatoire devant le conseil de prud'hommes pour rompre le contrat d'apprentissage peut constituer un frein à l'embauche pour les entreprises. Il peut aussi être éprouvant pour de jeunes apprentis, dont la période d'apprentissage est une première expérience du monde professionnel. En outre, la commission a renforcé le rôle du médiateur consulaire en cas de rupture du contrat sur l'initiative de l'employeur, afin d'assurer

Le cas de force majeure constitue un événement extérieur et imprévisible rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail. La rupture du contrat pour force majeure est prévue pour les CDD et les CDI.

7 rectifié. Licencier l'apprenti pour motif économique apparaît peu opportun et pas forcément nécessaire, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, la durée de l'apprentissage est assez courte : entre six mois et trois Deuxièmement, les employeurs sont exonérés de la quasi-totalité des charges patronales lors de l'emploi de l'apprenti : le salaire brut de l'apprenti est presque égal à son salaire net pour l'entreprise. Faciliter ainsi le licenciement de l'apprenti risquerait donc de fragiliser son statut de manière excessive. En revanche, rien n'interdit d'explorer une piste, avec le CFA, de reconversion dans une autre entreprise s'il n'y a plus la capacité de le former. En outre, un apprenti

Enfin, le versement de dommages et intérêts en cas de rupture anticipée du contrat n'apparaît pas opportun s'agissant de l'apprentissage. L'apprenti effectue une formation initiale et n'est pas dans un cas de précarité similaire à celui du bénéficiaire d'un CDD qui connaîtrait une rupture anticipée de son contrat. En cas de rupture sur l'initiative de l'apprenti, il apparaît compliqué d'exiger de celui-ci qu'il verse à l'entreprise des dommages et intérêts compte tenu de sa rémunération,

à l'instar de ce qui existe pour les CDD. Je suis favorable à cette proposition. Néanmoins, dans cette hypothèse, il conviendra évidemment de prévoir le régime indemnitaire dû en cas de rupture anticipée du contrat en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure.

Je suis évidemment favorable au fait de donner un plus grand rôle aux régions en matière d'orientation, car elles ont une vision transversale de la formation et de l'emploi dans leur territoire.

et les professions, ou DRONISEP, aux régions tout en voulant conserver l'Office est pour moi symptomatique d'une réforme qui ne va pas jusqu'au bout des choses. En effet, les DRONISEP sont les pompes à information de l'ONISEP. Les supprimer, c'est asphyxier l'Office. Le projet de loi porte donc en germe un ONISEP en apesanteur, coupé des territoires et des réalités du terrain. Le « mais en même temps » trouve donc ses limites.

et à tous ceux qui ont justement besoin d'un autre lieu que l'établissement scolaire pour construire un projet professionnel, une orientation fondée sur un autre regard que celui de l'école. Je suis aussi convaincu de leur rôle pour la coordination de l'action des psychologues de l'éducation nationale. En effet, nommer ces personnels en établissement va peut-être les rapprocher des élèves, mais aussi les isoler professionnellement. S'ils pouvaient jusqu'à présent développer un autre point de vue sur les élèves, c'était surtout parce qu'ils s'inscrivaient dans un autre collectif que l'établissement. Une régionalisation mal achevée, des CIO au lycée dans l'incertitude, des psychologues

en ce qui concerne les carrières liées au numérique. Le numérique sous-tend une mutation très profonde de notre société et de l'activité. Plus généralement, ce sont tous les métiers qui sont bouleversés par l'émergence de nouvelles compétences. de nouvelles compétences. Il faut une communication et une sensibilisation particulières auprès des jeunes filles pour qu'elles trouvent toute leur place dans les filières numériques. La proportion relative d'hommes et de femmes dans les métiers du numérique s'est fortement dégradée avec le temps dans notre pays. Alors que, en en 1972, l'informatique était la deuxième filière comportant le plus d'ingénieurs femmes, désormais, seuls 12 % des filles choisissent la filière de l'ingénierie numérique, ce qui a pour conséquence une masculinisation massive de ces métiers. À l'heure actuelle, seuls 6 % des développeurs sont des femmes ! Or la mixité est un enjeu important non seulement pour les individus- notamment en matière de lutte contre les inégalités salariales, qui sont souvent liées à la ségrégation des métiers par genre -, mais également pour les entreprises, en élargissant le vivier de recrutement et en leur permettant d'attirer de nouveaux talents. Plusieurs facteurs expliquent la faible attractivité du numérique auprès des femmes : d'une part, une image de la société fortement sexuée, qui enferme dès l'enfance filles et garçons dans des rôles déterminés à l'avance et qui se traduit par une vision « genrée » des métiers du numérique, renforcée par l'absence de modèle féminin part, une méconnaissance des métiers du numérique et de leurs finalités, alors que les choix d'orientation des filles sont moins déterminés par une appétence pour un métier spécifique que par un centre d'intérêt ou l'apport que les lycéennes souhaitent fournir à la société.

Certes, les dispositifs actuels sont perfectibles et nos jeunes méritent un accompagnement à la hauteur des enjeux qu'ils rencontrent pour se projeter et entamer sereinement leur vie étudiante et professionnelle. Pour autant, la remise en cause de la présence des CIO sur notre territoire ne me paraît pas un bon signal. Dans mon département des Pyrénées-Atlantiques, cinq centres réalisent un travail de proximité

qui divise nos territoires et n'offre pas les mêmes chances à chaque élève. La fracture numérique crée des inégalités considérables auxquelles les CIO peuvent répondre en accompagnant les familles les plus fragiles et non connectées. Alors, oui, faisons évoluer les CIO ! Réfléchissons à une meilleure articulation, révisons leurs objectifs et leurs missions, mais continuons d'assurer un maillage du territoire

Je tiens à rappeler les bienfaits du programme de rénovation de l'apprentissage que nous avons défini aux articles 7, 8 et 9

aux régions. Pour découvrir les métiers, pour diffuser l'information, la documentation, le projet professionnel, l'orientation des élèves et des familles, notre commission a renforcé le rôle des régions, ce qui est tout à fait normal.

deux branches : une branche dédiée aux actifs et sous la responsabilité des régions, l'autre restant sous l'autorité de l'État et destinée aux élèves et aux étudiants. Le transfert de la compétence d'information des élèves et étudiants aux régions questions, notamment sur la qualité de l'information dispensée, la qualification des personnes qui feront ces interventions et le contrôle des organismes mandatés par les régions.

cela reviendrait à priver le public scolaire du seul réseau public de proximité clairement identifié par les familles et dédié aux conseils sur la scolarité et l'orientation. C'est d'autant plus important que les personnels des CIO nous ont

En ce sens, cette fermeture annoncée, de même que le transfert du personnel des directions régionales de l'ONISEP aux régions, provoque à juste titre une très forte inquiétude chez les parents d'élèves.

Magner, pour présenter l'amendement n° 285 rectifié. Cet amendement vise à supprimer l'article 10 qui procède au transfert aux régions de l'organisation de l'information sur les métiers et les formations en direction des élèves et des étudiants, notamment dans les établissements scolaires. Notons d'abord qu'une telle disposition dans un projet de loi sur la formation professionnelle est à la limite de constituer un cavalier législatif ; je l'affirme en présence de M. le ministre de l'éducation nationale. Comment ne pas s'inquiéter des disparités dans les informations mises à la disposition des jeunes selon qu'ils habiteront dans tel ou tel territoire ? Comment ne pas s'inquiéter du poids que prendront les contraintes économiques locales et les entreprises locales dans les informations qui seront mises en avant par certaines régions ? Les informations sur l'orientation, aujourd'hui sous tutelle de l'État,

Sur les détails, je crains que le dispositif ne construise une véritable usine à gaz : les régions acquièrent cette nouvelle compétence, alors que l'État gardera la maîtrise de la définition de la politique nationale. cela s'apparente à une coquille vide ! Que pourra définir l'État, alors qu'il ne maîtrisera plus les modalités de transmission aux jeunes de sa politique d'orientation à l'échelon régional ? Par ailleurs, la majorité sénatoriale a aggravé le dispositif en supprimant les CIO, ce qui transparaissait déjà dans le dispositif initial. Les psychologues de l'éducation nationale seront donc contraints d'exercer uniquement dans les établissements scolaires et non plus dans ces centres où les élèves et leurs familles étaient habitués à venir les consulter dans un cadre tout à fait neutre. Que dire du transfert des personnels de l'ONISEP ? Sur quelles bases et selon quelles modalités s'effectuera-t-il ? Quant à la compensation financière prévue pour les régions, espérons qu'elle sera effective.

tous des améliorations. Nous en avons débattu en commission : l'article 10 renforce le rôle des régions en matière d'informations sur les métiers et les formations à destination des élèves et de leurs familles, ainsi que des étudiants. La connaissance par les régions des bassins d'emploi et leurs compétences en matière de développement économique leur permettra de fédérer les acteurs économiques sur tous les territoires régionaux au service d'actions d'information proches du milieu professionnel. Pour autant, à la lecture de l'article, la compétence de l'État en matière d'orientation et d'affectation des élèves et des étudiants n'est pas remise en cause. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

et je serais surpris que le Sénat qui, ici même, dans différents débats, nous soupçonne très souvent de vouloir donner trop de poids à l'État par rapport aux collectivités s'en offusque.

travaillent avec les régions pour de l'information de nature locale en lien avec un ONISEP qui garantit le caractère national de l'information et de la vision stratégique d'ensemble des enjeux d'orientation

Ce n'est faire offense à personne que de le dire, me semble-t-il : il y a aujourd'hui d'immenses frustrations en matière d'orientation, que ce soit de la part des personnels d'orientation, des élèves ou des familles. Il serait très hypocrite de faire comme si nous ne le savions pas. Dans ce contexte,

C'est exactement ce qui s'est passé cette année en classe de terminale : un second professeur principal a été nommé pour aider les élèves à s'orienter et cela s'est extrêmement bien passé. Dans ce contexte,

qu'attendent tous ceux qui, quoi que vous en pensiez, considèrent que l'on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui de l'orientation telle qu'elle est organisée dans notre pays et qu'il y a là un grand chantier à ouvrir. Au contraire, la loi ORE s'est malheureusement résumée de l'affectation le dispositif Parcoursup, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est ni le lieu ni le moment. Je ne m'attarderai pas sur l'avenir des CIO, qui nous inquiète beaucoup en termes de maillage territorial, mes collègues l'ont dit,

républicaine. Confier le travail d'orientation aux régions, au moment où notre société vit la mondialisation,

inquiets. Les messages très contradictoires qui sont envoyés aujourd'hui montrent que l'architecture globale de l'ONISEP et de ses délégations régionales

dès que l'on n'est pas d'accord avec vous, c'est forcément que l'on est mal intentionné, que l'on a mal compris, que l'on est de mauvaise foi. Pourtant, il ne me semble pas que vous déteniez seul la vérité, même si vous faites semblant de croire

en démembrant et en saucissonnant un service qui doit prendre l'enfant dans sa globalité, essayer de comprendre qui il est,

doit être une compétence partagée entre l'État et les régions. Concrètement, il s'agit d'inscrire dans la loi ce qui se fait en pratique,

Dans les deux cas, on risque de faire face à une catastrophe sociale de grande ampleur, à la fois pour les personnels, dont les postes sont en jeu, et pour les régions.

transfert aux régions de la compétence en matière d'orientation -aura pour première conséquence de faire disparaître un lieu d'exercice et de travail en équipe pour les psychologues de l'éducation nationale. Le projet global, qui consiste à transférer ces missions de conseil aux

Les CIO sont importants. Ce sont des lieux d'accueil ouverts toute l'année, qui couvrent un large territoire et qui apportent une aide au quotidien aux jeunes scolarisés, aux jeunes à besoins éducatifs particuliers, mais aussi aux élèves en situation de de décrochage scolaire ou encore aux adultes en reconversion professionnelle. Il est pour moi crucial de maintenir ces services publics de proximité dans nos territoires, sous la tutelle de l'éducation nationale. L'État doit conserver la responsabilité d'apporter une information fiable, neutre et gratuite. Il lui appartient de prendre en charge l'accompagnement

des territoires ruraux et offrirait à des officines privées, déjà bien implantées dans certains territoires, la possibilité de prendre le relais, privant les familles modestes de l'accompagnement dont elles bénéficiaient jusqu'alors.

est à M. le ministre. Cet amendement vise à rétablir l'article L. 313-4 du code de l'éducation, qui a été abrogé lors des travaux en commission. Cet article prévoit qu'est organisé dans chaque département un centre public d'orientation scolaire et professionnelle. Le Gouvernement ne souhaite pas remettre en cause cette obligation,

à prévoir une compétence conjointe entre la région et l'État pour l'organisation des actions d'information sur les métiers et les formations, contrairement à l'article 10, qui confie utilement cette compétence aux régions. La commission y est donc défavorable. tend à maintenir la présence d'un CIO dans chaque département et revient sur le principe de l'affectation des psychologues de l'éducation nationale dans les seuls établissements. Or la commission a considéré qu'il fallait enclencher la réorganisation des CIO et acter l'affectation des psychologues de l'éducation nationale dans les établissements. Ces mesures sont cohérentes avec l'expérimentation inscrite dans cet article, qui prévoit que ces personnels pourront être mis à disposition des régions.

Nous ne demandons pas de les faire disparaître, mais nous ne jugeons pas utile que le Gouvernement prévoie un article pour les maintenir. Nous préférons qu'il ait les mains libres pour sa réorganisation des services d'orientation, laquelle est absolument

qui se limiterait à organiser des actions d'information sur les métiers et les formations, mais bien une collectivité de plein exercice chargée de définir la politique d'information sur les métiers et les formations de son territoire. Cette rédaction traduit une approche

Les chambres consulaires contribuent à nourrir un réseau d'échanges entre acteurs économiques, entreprises, services publics et jeunes apprentis. Il convient donc de les associer aux actions d'information de la région.

confie aux régions des responsabilités en matière économique. Le présent amendement vise à prévoir, d'une part, que cette organisation se fait en lien avec les entreprises du territoire de la région, cette dernière étant la plus à même de les connaître, et, d'autre part, que les enseignants en charge de l'orientation sont également concernés par ces actions d'information.

rectifié visent à unifier les formulations figurant à l'article du code du travail qui définit les compétences de l'État et de la région en matière d'orientation. Ils sont donc de nature à clarifier les prérogatives partagées entre l'État et les régions

les articles 7 et 11 renforcent le rôle des chambres consulaires en matière d'apprentissage afin d'accompagner les entreprises dans l'embauche des apprentis, de former les maîtres d'apprentissage ou encore de réaliser certaines missions pour le compte des Les actions d'information sur les métiers et les formations confiées à la région pourront, si la région le souhaite, être réalisées avec des partenaires tels que des entreprises ou des chambres consulaires, à l'occasion par exemple de forums des métiers. conséquent, il n'est pas nécessaire de faire figurer cette précision dans la loi. Les partenaires des territoires doivent pouvoir passer des conventions et s'organiser en fonction des nécessités territoriales sans y être obligés par la loi.

qui définit un partage clair des missions entre l'État et la région. Il revient en effet à l'État de définir à l'échelon national la politique d'orientation des élèves et des étudiants. Celui-ci prend les décisions d'orientation et affecte les élèves. Il assume également la dimension éducative et pédagogique de l'orientation et de l'affectation des élèves, qui relève de ses missions de service public de l'éducation. La compétence d'information sur les métiers et les formations dévolue à la région n'est pas de même nature. Elle s'inscrit en complémentarité avec le rôle de l'État.